de plus de vingt-cinq ans dans 23 % des cas. De plus, les éléments de confort différaient entre les établissements publics et privés : si les Ehpad privés offraient quasiment exclusivement des chambres individuelles avec sanitaires privatifs, 11 % des places en Ehpad

L'article 16 reprend les dispositions actuelles donnant à la CNSA la compétence de contribuer au financement de l'habitat inclusif. Ce financement prend aujourd'hui la forme du forfait pour l'habitat inclusif, attribué à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée. La CNSA doit également pouvoir accompagner les initiatives des conseils départementaux et des métropoles dans leurs responsabilités de transformation de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat pour les personnes vulnérables. Elle doit même pouvoir évoluer vers le pilotage d'une politique de l'habitat en leur faveur, comme le suggère le rapport de Denis

Je rejoins votre souhait de poursuive le développement de cette nouvelle forme d'habitat, qui a initié un profond changement de perspective. Désormais, la lutte contre l'isolement, la pluralité de l'offre et, surtout, le maintien du lien social sont des outils à part entière de la prévention de la perte d'autonomie. nombreux porteurs de projets et acteurs institutionnels sont prêts. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis de sagesse sur cet amendement. De façon complémentaire, l'amendement gouvernemental n° 601, sur lequel la commission des affaires sociales a émis un avis favorable, vise à déployer dès le 1 janvier le dispositif proposé dans le rapport de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom. Je vous remercie,

l'avis du Gouvernement ? Cet amendement vise à modifier certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles pour les mettre en cohérence avec la nouvelle codification mise en place à l'article 16 du PLFSS. Je rappelle qu'une disposition habilitant le Gouvernement à prendre une ordonnance a précisément été prévue à cet effet. Elle a vocation à basculer les dispositions relatives à la CNSA du code de l'action sociale et des familles vers le code de la sécurité sociale. La codification sera réalisée à droit constant. Cette ordonnance permettra aussi de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux caisses nationales du régime général de la sécurité sociale au sein d'un même code, à savoir le code de la sécurité sociale.

l'amendement n° 130 rectifié. Cet amendement vise à financer la branche autonomie de la sécurité sociale en rehaussant la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA). Le doublement de cette contribution permettra d'abonder la branche de près de 3 milliards d'euros. En conséquence, davantage d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prévues par cette cinquième branche pourront être financées. La branche autonomie, créée à l'été 2020, ne bénéficie pas de financement pérenne, mais d'un simple redéploiement de crédit. Le rapport Libault a mis en avant le fait que 10 milliards d'euros annuels seraient nécessaires pour financer correctement la dépendance et la perte d'autonomie. Cet amendement vise donc à pérenniser les financements de la branche autonomie de la sécurité sociale en remplaçant, de manière strictement proportionnelle, une partie de la fraction de CSG allouée au financement des recettes de la CNSA. À ce jour, la CSA À ce jour, la CSA est due dans le cadre de la « journée de solidarité », journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Elle rapporte près de 3 milliards d'euros annuels. En 2020, la journée de solidarité devrait permettre de collecter 2,948 milliards d'euros au profit de la CNSA. Le doublement de la CSA

Le groupe CRCE propose depuis des années qu'une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie prise sur les revenus des actionnaires et de la finance soit mise en place. Une telle mesure contribuerait à faire de l'autonomie un enjeu de société. Le principe des quatre branches de la sécurité sociale

? Relever le taux de la CSA aurait pour effet d'augmenter la contribution des employeurs, ce qui se traduira automatiquement par une augmentation du coût du travail.

majoritairement des personnes âgées. Cela pourrait rapporter près de 3 milliards d'euros à la branche et contribuer ainsi, en partie seulement, à répondre aux besoins.

d'une maison solide et qui tiendra longtemps. Monsieur Milon, le texte n'est pas totalement dénué de sens, puisque, d'une part, un certain nombre de vos amendements

dilatoire. Rien n'empêcherait de voter des recettes et de continuer le chemin pour améliorer le dispositif, même si- cela a été dit précédemment -on a complètement inversé la donne.

pour des raisons idéologiques. C'est ça, la réalité

rectifié. Il s'agit d'un sujet sensible. Aux termes de l'article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la cinquième branche de la sécurité sociale consacrée au financement de la politique de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Plus précisément, cet article prévoit que la CNSA gère un nombre limité d'enveloppes, sans recettes affectées, correspondant à de grandes catégories de dépenses. Celles-ci recouvrent la totalité des dépenses actuellement dans le périmètre de la CNSA, dont l'OGD, l'objectif global de dépenses, et les concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), mais également l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est une prestation en espèces de la branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé [ ...], si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. « Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Afin de faire évoluer cette prestation, l'IGAS a été chargée d'une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l'objectif premier était d'aboutir à une « évolution de l'AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation mission, remis par Daniel Lenoir en juin 2019, identifiait les problématiques et proposait des scénarios, qui n'ont pas fait l'objet de concertations à ce stade. Le rapport de Laurent Vachey préconise le transfert de l'AEEH à la branche autonomie, ce que traduit cet article, qui acte ce transfert et le motive, dans le dossier de presse, par le fait que cela permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ». Or l'AEEH constitue une allocation familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l'allocation de soutien familial permet de prendre en compte le fait d'être un parent isolé ou que l'allocation de rentrée scolaire permet de tenir compte Certains éléments des compléments de l'AEEH relèvent néanmoins de besoins de compensation- aides humaines ou techniques, frais spécifiques ou autres -, quand d'autres permettent à un parent de réduire ou de cesser son activité professionnelle de s'occuper de l'enfant ou d'avoir recours à l'embauche d'une tierce personne rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH Enfant. Néanmoins, cela ne pourrait se faire qu'après les concertations attendues depuis la remise de rapport de l'IGAS. C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer les alinéas organisant ce transfert, afin de repousser cette décision au terme des concertations qui décideront d'intégrer l'AEEH, en tout ou partie, au travers de l'ordonnance prévue par le III de l'article visé. Cette suppression doit s'accompagner de l'engagement du Gouvernement à entamer des concertations sur le sujet. La

nécessite une concertation préalable avec les familles et les associations intervenant dans le champ du handicap, qui n'a pas eu lieu pour l'instant. En effet, la compensation des charges et la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs de la politique familiale. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vise à compenser les dépenses liées à une situation de handicap d'un enfant et les pertes de salaires subies par les parents, qui sont bien souvent dans l'obligation de réduire leur activité professionnelle.

? Si l'on suivait cette logique jusqu'au bout, ce serait l'ensemble des dépenses liées au handicap et intégrées dans le champ des prestations familiales qui devrait alors être pris en charge par la branche autonomie.

allocation dans le périmètre des prestations familiales garantirait aux familles une équité de traitement sur l'ensemble du territoire, contrairement à ce qui est parfois reproché aux MDPH. J'insiste en outre sur la nécessité d'une concertation avec les familles de personnes handicapées.

du 15 décembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées avaient chargé l'IGAS d'une mission relative à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l'objectif premier était d'aboutir à une « évolution de l'AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation

doivent faire, selon nous, l'objet de concertation et de travaux préalables en 2021, afin de vérifier et de justifier de la pertinence d'un transfert partiel ou total vers la branche autonomie. En d'autres termes, il est urgent d'attendre. Nous demandons un peu de patience avant de prendre une telle décision de transfert, qui nous semble, ainsi qu'aux acteurs du handicap, tout à fait prématurée.

visent à supprimer l'intégration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au sein du périmètre de la branche autonomie. Cette allocation, parce qu'elle s'adresse aux familles dont l'un des enfants est handicapé, se trouve naturellement, dans l'esprit de beaucoup, à la frontière entre la branche famille et la branche autonomie. La prestation de compensation du handicap, elle, est bien une prestation de compensation par nature, donc elle est attachée à la branche autonomie. Dès lors, pour nous donner les moyens d'articuler ces deux prestations, déjà liées, d'ailleurs, par un droit d'option, droit d'option, très complexe pour les familles, nous les avons rapprochées au sein de la cinquième branche. Je dis bien « rapprochées » et non pas « fondues », car les logiques de prestation familiale et de compensation du handicap ont une nature différente, et les acteurs sont particulièrement attachés à cette distinction. les sénateurs, ainsi que les associations, l'allocation de base de l'AEEH conserve ses mécanismes et ses critères d'attribution ; elle est bien instruite par les MDPH,

en cohérence avec le code de la sécurité sociale. Une telle habilitation est d'autant moins nécessaire que le Gouvernement nous annonce l'examen imminent d'une grande réforme de la prise en charge de la perte d'autonomie. Il paraît donc naturel

Je vais ajouter un argument à ce que vient de dire M. Milon.

précisé que « le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi,

la loi sur le grand âge et l'autonomie. Il n'y a donc pas besoin d'ordonnances ; nous voterons la loi directement. Faites un peu confiance au Parlement, il sait travailler rapidement, pour peu que le Gouvernement le saisisse.

codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévues au code de l'action sociale et des familles ». Monsieur le rapporteur général, il s'agit là de mesures de légistique,

Cet amendement tend à confirmer le rôle de partenaire de la CNSA et d'acteur de la mise en oeuvre de la cinquième branche sur les territoires que joue le réseau des caisses de MSA. Une convention avec la CNSA précisera le cadre de ce partenariat. Quel est l'avis du Gouvernement

les salariés et les non-salariés agricoles. La CNSA, chargée de la gestion de la branche autonomie depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie, a ainsi vocation à agir comme aujourd'hui pour l'ensemble des personnes âgées et des personnes handicapées, qui sont toutes rattachées au régime général pour la couverture de ce risque. L'amendement que vous nous proposez, monsieur le rapporteur général, aboutirait, nous semble-t-il, à remettre en cause la visée universaliste de la nouvelle branche. Il aurait ainsi pour effet de complexifier par avance le pilotage de la politique en matière d'autonomie.

Alors que la France est parfois hâtivement dépeinte comme le lieu du conflit social permanent et d'une étatisation excessive- quand ce n'est pas prédatrice -, il s'avère que notre pays a confié près d'un quart de sa protection sociale, 150 milliards d'euros, aux représentants des salariés et des employeurs parce qu'ils semblaient les mieux à même de s'occuper de certains sujets touchant à la vie de tous les jours, pour le salarié et sa famille : les retraites complémentaires, le chômage, la prévoyance, la santé au travail, la formation professionnelle, le logement ou l'insertion des personnes handicapées sont aujourd'hui l'affaire des partenaires sociaux au moins autant que de l'État précise également que, « partout où les partenaires sociaux se sont vu confier ou se sont saisis de véritables responsabilités, cette confiance dans des corps intermédiaires pourtant très critiqués s'est traduite par une gestion consensuelle et sérieuse des cotisations des salariés et des employeurs La création d'une cinquième branche de la sécurité sociale ne peut, de fait, se concevoir sans la mise en place d'une organisation paritaire, sauf à retomber dans une logique jacobine centralisatrice sur cet enjeu majeur pour la société française, ce qui serait le meilleur moyen de fragiliser encore davantage notre modèle social. La société française souffre d'un légitime sentiment de dépossession de son pouvoir de décision et de sa souveraineté sur les questions qui la concernent au premier chef. Nous n'avons pas les moyens de continuer à la fracturer en minorant le rôle des partenaires sociaux dans la gestion de la cinquième branche de la sécurité sociale qu'est destinée à devenir la branche autonomie ni à faire l'économie de la négociation collective sur les enjeux majeurs de notre temps. La construction de la cinquième branche nécessite un travail de concertation sérieux et de longue haleine, concentré sur le paritarisme, d'autant plus que « le fait que des représentants des salariés et des employeurs, comptés en nombre égal, se réunissent pour créer de la norme, pour l'interpréter et pour gérer les institutions et les droits qui en sont issus est un procédé aussi simple à comprendre que difficile à mettre en oeuvre ». La loi doit prévoir les modalités de la mise en place du paritarisme au sein de la branche autonomie de la sécurité sociale. Tel est l'objet du présent amendement. Quel est l'avis

En France, 7 436 établissements d'hébergement accueillent à peu près 605 000 personnes âgées dépendantes. Il se trouve qu'un certain nombre de ces établissements pratiquent la fraude et l'évasion fiscales de façon absolument remarquable.

le PLFSS donne des moyens à cette nouvelle branche, afin qu'elle puisse justement ne pas rester cette coquille vide tant critiquée. Les débats continuent d'enrichir la cinquième branche. Les échanges en première lecture à l'Assemblée nationale l'ont démontré. La CNSA aura désormais, par exemple, la mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des personnes exerçant les métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes atteintes de handicap

que sur les engagements du Gouvernement. Si, pour agir, nous attendons que toutes les mains se lèvent, nous attendrons longtemps ! Avec ce PLFSS, la cinquième branche se dessine. Les missions de la CNSA sont essentielles pour répondre aux besoins de tant de citoyens. Nous saluons cet article, que nous voterons. Il représente l'action, il marque une amélioration pour de nombreux citoyens et, surtout, engage l'avenir. Nous nous en félicitons. La

Ils attendent une vision globale de l'avenir pour notre vieillesse. Cette question est source d'angoisse pour la société française, qui sait que c'est l'un des grands défis qu'elle devra relever. On ne règle rien sur le fond. On ne règle rien stratégiquement. On ne règle rien financièrement. On croit qu'un effet d'annonce suffira à convaincre l'opinion,

Madame la sénatrice,

de passer à la définition des financements, des contenus et du mode de gestion de ce qui se doit d'être un progrès social, à savoir la gestion par la sécurité sociale du risque autonomie.

Tout doit être mis sur la table : raison pour laquelle nous voterons cet article 16.

Le scrutin est ouvert.

concernant un projet de loi Grand âge et autonomie en 2021, mais le Sénat souhaite marquer de son empreinte ce rendez-vous sur le débat financier. donc à réunir une conférence des financeurs de la politique de soutien à l'autonomie, sous l'égide de la CNSA, pour faire des propositions relatives aux financements nouveaux nouveaux que requiert l'organisation par la branche autonomie et les collectivités territoriales d'une prise en charge des personnes en perte d'autonomie privilégiant le maintien à domicile. La promesse d'une grande réforme de la dépendance à fêter son deuxième anniversaire récemment, puisque la constatation Grand âge et autonomie a été lancée le 1 octobre 2018. Depuis, des travaux utiles ont été publiés, mais peu de mesures concrètes ont été décidées, en particulier sur la délicate question du financement d'une meilleure prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, c'est-à-dire d'un virage domiciliaire. Cet amendement vise à catalyser la prise de décision ou, au moins, à maintenir le sujet à l'agenda politique. Quel est l'avis du Gouvernement

l'amendement n° 724 rectifié. Au début de l'examen de l'article 16, j'ai souligné la nécessité que cette cinquième branche réponde à la demande d'universalité qu'exigent les personnes en perte d'autonomie. Tout doit être mis en oeuvre pour faire converger les politiques de l'âge et du handicap.

ou après 60 ans, les personnes ont accès soit à la prestation compensatoire du handicap, soit à l'allocation personnalisée d'autonomie versée aux personnes âgées dépendantes. Ces deux prestations sont d'une nature et d'un montant différents. Le secteur associatif du handicap estime que le chantier de la cinquième branche doit permettre d'abroger définitivement « la barrière d'âge des 60 ans » et rappelle qu'il est temps de réduire le morcellement des dispositifs et de sortir de la logique de catégorisation des publics.

qu'il s'agit d'une personne âgée ou d'un enfant en devenir d'autonomie. Nous ouvrons aussi plus largement les droits à compensation aux personnes les plus âgées avec l'ouverture du droit à la PCH au-delà de 75 ans pour les personnes répondant aux critères d'éligibilité de la PCH avant 60 ans. L'heure est

Le récent rapport de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom montre que l'essor de ces formules de plus en plus plébiscitées appelle un financement plus fluide de la fonction d'animation du lieu de vie. Il propose ainsi d'instaurer une aide à la vie partagée, octroyée à tout habitant d'un habitat inclusif dont le bailleur ou l'association gestionnaire a passé pour cet habitat une convention avec le département. Cet amendement vise à permettre la mise en oeuvre de cette aide à la vie partagée dans le règlement départemental d'action sociale en assurant une couverture partagée de son coût entre le département, signataire de la convention, et la CNSA. Pour donner une impulsion forte, la CNSA garantira la couverture de tout ou partie des conventions signées par les départements avant fin 2022 à un taux d'au moins 80 %. Le montant prévisionnel atteindra 20 millions d'euros dès 2022, ce qui correspond au financement d'environ 500 projets de cinq à dix logements sur l'ensemble du territoire. La création de cette aide à la vie partagée permettra de mener sur

l'avis de la commission ? Cet amendement vise à autoriser les règlements départementaux d'aide sociale à prévoir une aide à la vie partagée à l'attention des habitants d'une formule d'habitat inclusif dont le financement serait coassuré par la CNSA à hauteur de 80

de la taxe sur les salaires, comme cela se fait déjà pour l'État et les collectivités territoriales. Alors que les personnels hospitaliers réclament de nouveaux moyens financiers et humains d'ampleur, cette mesure permettrait de déployer 5 milliards d'euros dans l'activité hospitalière dès 2020. Certains nous opposeront que, si les hôpitaux et les Ehpad publics paient une taxe sur les salaires, c'est parce qu'ils ne sont pas astreints à payer la TVA. Mais je peux vous citer des établissements publics qui ne sont pas astreints à payer la TVA et qui sont exonérés de la taxe sur les salaires. Je pense notamment aux collectivités locales et à leurs régies, aux centres d'action sociale, aux centres de formation des personnels communaux, aux établissements d'enseignement supérieur. Finalement, seuls les hôpitaux

de l'exonération de la taxe sur les salaires, par le biais du CITS. On peut donc considérer qu'il existe actuellement une situation déloyale à l'encontre des hôpitaux et des Ehpad publics.

est étonnant de constater que ce débat a lieu en réponse à notre proposition, alors qu'il n'a jamais eu lieu lors de la création du CICE, du CITS, du CIR et autres exonérations de cotisations.

Dans le cadre des réflexions qui se font jour concernant la prise en charge du grand âge, il convient de lutter contre les restes à charge astronomiques des résidents des Ehpad. Comme l'observe le rapport de mars 2018 des députées Iborra et Fiat, une telle évolution nécessite de transférer certains postes, aujourd'hui financés

Nous constatons que, si nous étions peu nombreux au départ, la multiplication des pénuries de médicaments et la crise sanitaire de la covid-19 ont convaincu de nombreuses associations, des professionnels de santé et des citoyennes et citoyens que l'État devait reprendre la main. L'État ne peut plus rester sans rien faire et dépendre des stratégies des laboratoires, qui ont délocalisé la production de médicaments vers les pays d'Asie. Je pense également aux comportements de certains grossistes-répartiteurs, qui préfèrent vendre leurs stocks de médicaments aux pays les plus offrants, ainsi qu'aux tensions sur les approvisionnements, volontairement créées par les laboratoires pour faire augmenter les prix. Les autorités publiques sont sommées d'agir pour garantir un service essentiel, à savoir l'accès universel aux soins de santé et aux médicaments. Pour rappel, en 2019, ce sont plus de 1 200 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui ont été concernés par des tensions ou une rupture d'approvisionnement, contre 800 en 2018. L'obligation pour les industriels de constituer un stock de sécurité votée l'an dernier était un premier pas- je reviendrai sur les lacunes du dispositif, en particulier sur le décret du ministre de la santé limitant à deux mois la couverture des besoins en médicaments.

Sachant que le contexte sanitaire doit nous amener à réfléchir dans les mois à venir sur le choix du mode de production du futur vaccin contre la covid-19, nous proposerons, dans le cadre de ce débat, une production publique du vaccin permettant de garantir le respect des meilleures conditions de sécurité et de transparence, ainsi qu'un tarif ne créant pas une dépense excessive pour la sécurité sociale. En réalité, nous voulons que ce vaccin soit accessible à toutes et tous sur l'ensemble de la planète, qu'il soit gratuit et, pour ce qui concerne la France, qu'il soit remboursé à 100 % par la sécurité sociale.

La commission des affaires sociales a débattu de plusieurs amendements portant sur quatre thèmes distincts, que les aléas de la discussion nous feront tour à tour aborder, mais qu'il convient de ne pas confondre. Premièrement : la clause de sauvegarde des médicaments. Il s'agit d'un mécanisme fiscal qui vise à juguler en dernier recours les dépenses d'assurance maladie en matière de médicaments et qui soulève depuis plusieurs années les contestations des acteurs pharmaceutiques.

Un amendement de nos collègues René-Paul Savary et Bruno Retailleau visera à prendre en compte les évolutions industrielles en matière de médicaments dans l'Union européenne.

des dépenses de santé. Le Gouvernement a donc aménagé la clause de sauvegarde, en minorant le taux d'abattement dont les laboratoires bénéficiaient jusqu'à présent, le faisant passer de 20 % à 5 %. Il est normal que les entreprises pharmaceutiques soient mises à contribution et s'impliquent dans la politique de baisse des prix des produits de santé menée par le CEPS. C'est pourquoi le Gouvernement leur offre la possibilité de s'acquitter de leur contribution par le biais d'une baisse du prix de leurs médicaments, avec cette fois-ci une fenêtre d'abattement Il n'en reste pas moins que la minoration de l'abattement de base à 5 % est grandement préjudiciable, non seulement pour les petites structures avec des moyens moins importants, mais également pour l'attractivité de notre territoire des investissements et des expérimentations cliniques dont tant de patients atteints de pathologies rares et lourdes ont besoin. À défaut de À défaut de trouver de meilleures solutions, il convient que ce nouveau mécanisme de pression à la baisse des prix soit incitatif pour les entreprises. Il doit être plus intéressant pour les laboratoires

pour toute entreprise ayant consenti à une baisse de son prix net de référence. Une telle individualisation de la négociation, bien qu'elle ait suscité la perplexité, puis les doutes, du secteur présente au moins, selon moi, l'intérêt de tenter

et de l'amélioration de la santé de nos patients. Les procédés actuels nécessitent énormément de recherches. Selon moi, le nivellement par le bas n'est pas la bonne solution.

est à Mme Annie Delmont-Koropoulis. La politique de négociation conventionnelle sur les prix entre le CEPS et les entreprises pharmaceutiques repose sur la confiance et la responsabilité de chaque partie. Chacune d'elle sait que le coût de l'innovation est justement évalué et qu'il permettra un accès équitable de chacun aux produits de santé. C'est d'ailleurs sur ce fondement que près de 95 % des laboratoires ont conventionné avec le CEPS. La relation contractuelle entre le CEPS et les entreprises pharmaceutiques a permis à la France d'être leader en matière de production de médicaments en Europe et d'être un important créateur d'emplois industriels, ce qui risque de ne plus être le cas désormais. Il est essentiel que la politique conventionnelle soit protégée et promue par le législateur. Les garanties apportées par cette méthode sont importantes pour que chaque patient puisse avoir accès à des stratégies thérapeutiques de qualité et, pour ceux

à un accord-cadre négocié entre le CEPS et les syndicats des entreprises pharmaceutiques plutôt qu'à un arrêté ministériel. Quel

Comme le rappelait voilà quelques jours l'association UFC-Que Choisir, les pénuries explosent : plus de 1 200 médicaments étaient concernés en 2019, et l'Agence nationale de sécurité du médicament prévoit le double pour 2020, notamment du fait de la crise sanitaire. Au-delà des ruptures, c'est la durée d'attente qui est inquiétante. En 2017, les usagers ont dû attendre en moyenne avant de constater un retour à la normale de l'approvisionnement de leurs médicaments. Les vaccins sont les plus touchés : ils sont en moyenne indisponibles pendant 179 jours, soit près de six mois.

vote. Ce que vous nous proposez, ma chère collègue, c'est une dérégulation : on retire à l'État sa capacité d'arbitrage. Je ne pense pas que l'État soit bête au point de tordre le cou des industries du médicament, en ne tenant absolument pas compte de leurs arguments. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre l'intérêt général et la production et l'innovation sur notre territoire.

qui n'a d'ailleurs qu'une existence facultative, est de normer le plus légèrement possible les négociations entre l'industriel et le CEPS au moment de la définition des remises. Il ne me paraît pas souhaitable d'y faire figurer un élément susceptible d'infléchir

du Gouvernement. Cette instance, vous le savez, a pour mission, fixée par la loi, de déterminer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge par l'assurance maladie. Il nous semble donc que les éléments supplémentaires que vous

Et la tarification fixée par le CEPS entre en ligne de compte dans les critères utilisés par ces entreprises pour décider si elles restent ou non en France.

un certain nombre de dispositions, d'ailleurs, se trouvent plutôt dans le projet de loi de finances que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette politique se trouve donc en différents endroits. me garderai bien de donner des conseils à la Haute Assemblée, mais elle dispose, me semble-t-il, d'un certain nombre d'instruments, d'outils, d'évaluation

il me semble qu'avec un peu d'ingéniosité, sans tomber dans le protectionnisme étroit, on pourrait quand même, du point de vue des remboursements, favoriser un juste prix pour ce qui est produit en France et être plus exigeant pour ce qui ne l'est pas. Or, paradoxalement, c'est plutôt l'inverse qui se passe : comme on nous dit que les autres pays ne veulent pas nous vendre à moins de nous vendre cher, nous acceptons de payer cher à l'importation

extrêmement important et urgent.

Dans ce contexte exceptionnel, le secteur de la répartition a fait preuve d'une mobilisation sans précédent pour répondre à l'ensemble des demandes des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, en assurant notamment, avec les pharmaciens, la distribution de plus de 600 millions de masques chirurgicaux et FFP2. Outre ces missions supplémentaires assurées tout au long de la crise, les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent au quotidien un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l'approvisionnement des 21 000 pharmacies françaises, sur l'ensemble du territoire.

les pertes de 2020 devraient être elles aussi significatives, alors que plusieurs entreprises ont déjà dû mettre en place des plans de sauvegarde de l'emploi. Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels de la répartition alertent sur la situation économique de leur secteur, qui s'aggrave chaque année et en est aujourd'hui à un point très critique. Ils Ils accumulent les pertes en raison d'une rémunération réglementée qui ne correspond plus aux coûts que le secteur doit supporter, à quoi s'ajoute, comme je le disais, un modèle fiscal antiéconomique et confiscatoire. Pourtant, des Pourtant, des discussions existent avec les pouvoirs publics depuis l'automne 2018 ; elles ont notamment permis de définir de nouvelles règles de rémunération, mais elles ne corrigent que très partiellement ces déséquilibres et laissent le secteur dans une situation de précarité.

Il s'agit du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires des grossistes-répartiteurs. Je rappelle qu'en 2018 ce chiffre d'affaires était à peu près de 17 milliards d'euros ; il se traduisait pour la profession par un excédent brut d'exploitation de 200 millions d'euros. Les grossistes-répartiteurs estiment aujourd'hui qu'un allégement du taux de cette fiscalité sur leur chiffre d'affaires à 1,4

Rappelons, vous l'avez fait, le rôle qu'ont joué les grossistes-répartiteurs dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Ils ont apporté leur contribution sur des missions exceptionnelles, comme la sénatrice Valérie Boyer, dont je salue l'arrivée au Sénat, le rappelait : la livraison des masques ou encore de certains médicaments aux officines, afin d'éviter les déplacements de patients. Ces missions ont donné lieu à des prises en charge spécifiques. Les missions relatives aux masques ont engendré, pour les

et officines. Afin de compenser leur baisse d'activité alors qu'ils subissent des coûts fixes, une mesure d'urgence de 30 millions d'euros a en outre été décidée, une revalorisation des marges, dans l'arrêté publié le mois dernier. Cette revalorisation s'appliquera dès le dernier trimestre de 2020. Ce montant a d'ores et déjà été pérennisé pour les années suivantes.

d'euros annuels, qui sont donc pérennisés, nous étudions différentes pistes pour rendre la marge de ces acteurs moins sensible à l'évolution du prix des médicaments, notamment par la mise en place d'une rémunération par forfait pour certaines missions importantes.

devaient cesser. Il faut respecter le Parlement

que celles proposées par les sénateurs, qui d'ailleurs n'imposent pas de passer par la loi, car tout ne passe pas forcément par la loi,

de la santé. J'en viens à mon amendement. L'article 17 précise le montant du taux Z pour 2021 concernant la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois, le dispositif mis en place à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ne prévoit pas de mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical, constitué en majorité de PME, TPE et ETI. Le présent amendement vise à intégrer

des médicaments, souligné dans l'exposé des motifs, est certes séduisant, mais nous fait oublier que, contrairement aux médicaments, la dynamique de dépenses des dispositifs médicaux est beaucoup plus importante et nettement supérieure au barème de l'Ondam. La Cour des comptes, dans son récent rapport, a souligné l'importance de ce sujet et nous a conviés à la plus grande vigilance.

de manière incidente -, de nombreux débats. Le Gouvernement avait émis un avis défavorable, et cet amendement avait été rejeté. Par souci peut-être de constance, l'avis du Gouvernement sera également défavorable cette année, pour des raisons de fond que je me permets d'exposer à

je partage avec vous la volonté d'engager avec le secteur des dispositifs médicaux des échanges un peu plus structurés que ceux que nous avions, encore aujourd'hui même,

que les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l'outil de production, dans l'Union européenne, le Royaume-Uni et en Suisse, ainsi que les étapes de fabrication des médicaments ou des dispositifs médicaux- il nous faut prévoir dès maintenant

la localisation de production en France peut aider à la sécurisation des approvisionnements, ce qui est, comme nous le voyons au cours de cette crise, un enjeu majeur. Votre amendement fait cependant un lien direct entre fixation du prix et implantation des entreprises en France. Une fois encore, la question de l'implantation des entreprises en France dépend de beaucoup d'autres leviers qu'actionne le Gouvernement : le financement des projets de recherche, le soutien des essais cliniques, le crédit d'impôt recherche, etc. L'enjeu des implantations nationales et de leur impact pour la sécurisation des approvisionnements sera travaillé dans l'accord-cadre en cours de négociation avec l'industrie. Le Gouvernement, pour toutes ces raisons, émet un avis défavorable.

Merci,